Monsieur le président,

la soirée, mon rappel au règlement concerne les modalités d'application de l'article 45 de la Constitution à l'occasion de l'examen de ce projet de loi. Cet article parfaitement limpide prévoit, dans son premier alinéa : « Sans préjudice des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect- cette expression -, avec le texte déposé ou transmis. » Limpide ? Apparemment pas pour tout le monde, puisque la commission des lois, à la sauvette, sans dire qui est à l'origine d'une telle décision, sans autre commentaire que le renvoi à l'article 45, a déclaré irrecevables sept amendements qui avaient pour objet la révision du code pénal, afin de mieux prendre en compte la situation et les obligations que les maires tiennent de leur mandat électif : définitions des notions de prise illégale d'intérêt, de favoritisme et du champ de l'irresponsabilité pénale. Elle a en outre retoqué sept autres amendements visant le conflit d'intérêts. Beau tableau de chasse ! Ce projet de loi comportant un titre intitulé « Renforcer et reconnaître les droits des élus », j'en conclus que pour la commission des lois du Sénat, lesdits élus n'ont pas d'autre droit que de se laisser insulter, taper sur la tête, renverser par des engins dans l'exercice de leurs fonctions en psalmodiant les douze « préconisations » lénifiantes publiées au nom de la commission, en en réponse aux menaces et agressions auxquelles ils sont confrontés. Certes, je n'ignore pas que le parlementarisme « rationalisé » est un parlementarisme avec une muselière. Je considère néanmoins que le bon toutou n'est pas obligé d'aimer cette muselière, encore moins de réclamer qu'elle soit la plus serrée possible. Il est grand temps, mes chers collègues, de faire cesser ces dérives, qui, en restreignant notre liberté d'amendement, minent la confiance des élus locaux dans notre capacité à les représenter et à les défendre et, par-delà, minent la légitimité du Sénat. Lors d'un entretien diffusé à la télévision il y

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, on peut se faire plaisir, mais on peut aussi faire oeuvre utile. Je suis très peu intervenu dans ce débat et j'ai assisté à presque toutes les séances consacrées à ce projet de loi, dont l'importance ne vous a pas échappé et dont l'utilité pour les élus locaux est réelle.

puisse rester facultative. Il s'agit ainsi de répondre aux difficultés rencontrées dans certaines communes nouvelles, qui ne trouvent pas assez de candidats au conseil municipal pour satisfaire cette obligation. J'ai notamment en tête l'exemple de la commune nouvelle de Porte-de-Benauge en Gironde, pour laquelle avoir entrepris cette démarche représente un cadeau empoisonné pour les prochaines municipales de mars 2020. Si la logique qui sous-tend l'article 1 du texte de loi a été d'encourager la fusion de communes, force est de constater que, au vu d'une relative désaffection des citoyens pour le mandat local, cette disposition a visée incitative peut aussi avoir l'effet inverse et créer une difficulté nouvelle pour la commune nouvelle.

car il est actuellement impossible de mutualiser les moyens humains et matériels entre les services de voirie, par exemple d'un département et d'une commune ou d'une intercommunalité, le code général des collectivités territoriales, le CGCT, ne le prévoyant pas. La transposition aux conseils départementaux de ces mécanismes de mutualisation des services déjà applicables applicables aux communes et EPCI pourrait offrir à ces collectivités l'opportunité de disposer d'un outil. Cette mutualisation présenterait un intérêt économique d'abord pour assurer l'entretien des réseaux routiers des collectivités, notamment rurales. Les possibilités de mutualisation des ressources en moyens matériels et humains pourraient permettre des performances accrues, au bénéfice tout particulièrement des EPCI fraîchement nés, non encore organisés, qui seraient efficacement aidés. Il s'agit de mettre en adéquation l'usage des moyens au regard des besoins à une échelle d'intervention complémentaire et pertinente, source bien évidemment d'économies budgétaires. Cela constituerait un outil supplémentaire facilitateur pour le développement des territoires,

aboutirait à un tout autre résultat, puisque l'on ajoute les départements à la liste des groupements de collectivités territoriales définis par le CGCT, alors que le département est aujourd'hui une collectivité territoriale à part entière. Je vous demande de retirer votre

à une demande très forte du département et des EPCI concernés.

aux parents le choix de déclaration du lieu de naissance de leur enfant. Ceux-ci pourraient déclarer la naissance soit auprès de l'état civil de la commune où l'enfant a effectivement vu le jour, soit auprès de celui de la localité de leur

dans le fait que plus aucun enfant ne sera déclaré né dans cette ville, qui est pourtant une préfecture. À la suite des restructurations territoriales de l'offre de soin, des sites d'accouchements ferment. Force est de constater que, dans les territoires ruraux, le lieu de naissance est parfois situé dans un autre département que

de ses parents.

La loi NOTRe a sacrifié les petites communautés de communes et les services de proximité au fil des années. Dans des communautés de communes comme la mienne, qui regroupe 68 communes sur un très grand territoire,

de notre collègue pour que nous nous rassemblions autour de la défense des territoires et de l'exercice de la compétence au bon niveau. Mon cher collègue, la semaine dernière, nous avons

Il est vital pour les territoires ruraux, la création des communautés de communes « XXL » ayant véritablement signifié une marche arrière terrible pour les petites communes sur les territoires ruraux.

certain nombre de conseils. Ainsi, de 2001 à 2015, les effectifs des services placés sous l'autorité des préfets ont perdu près de 10 000 emplois, soit une baisse de 11 %. la Cour des comptes, en 2017, regrettait que de nombreuses missions de l'État soient en situation de tension ou de risque, avec des missions délaissées ou mal exercées, comme le traitement des aides aux agriculteurs, au titre de la politique agricole commune, par la direction départementale des territoires

ce qui, de fait, pénalise les communes en termes de montant des aides qu'elles peuvent recevoir. Nous souhaitons regarder ce problème de plus près. Il nous paraît nécessaire de détailler les évolutions des moyens humains et financiers des services déconcentrés de l'État,

: « Le sentiment général est que la parole de l'élu rural n'est pas entendue et que le maire qui incarne la proximité se trouve trop souvent dépourvu face à des mesures de plus en plus complexes à appréhender. Un double sentiment de frustration se fait jour : l'incapacité d'expliquer à ses administrés les mesures prises au-delà de la commune et le sentiment d'être spectateurs plutôt que d'être des décideurs. Le sentiment d'impuissance chez les élus ruraux persiste. » Dans nos territoires, nous constatons tous que le désengagement des préfectures en matière d'ingénierie n'a pas été compensé de manière satisfaisante. Les autres échelons, notamment le département, ne comblent pas toujours totalement les besoins. Une évaluation régulière est manifestement nécessaire, en particulier pour le Sénat, qui doit être un garant de l'effectivité de l'exercice des compétences des collectivités territoriales.

d'identité, dans la mesure où de nombreuses communes ont vu leurs compétences en matière d'état civil fortement se réduire.

du Gouvernement de réaffirmer le rôle de la commune dans ce qui fait République, dans ce qui fait du commun et dans de ce qui fait la citoyenneté dans notre pays.

Les maires ruraux de votre département comme du mien ne connaissent plus leur population. Les administrés n'ont plus aucune raison, s'il n'y a pas d'école et qu'ils n'ont pas d'enfants scolarisés, de venir

on coupe complètement le lien entre les maires et leur population. Je sais que l'on peut aussi développer des services comme le dépôt postal. Très bien ! Certaines communes le font, mais La Poste ne le prévoit pas pour toutes.

Malheureusement, le respect de cette prise de position formelle par ladite collectivité locale a peu de conséquences juridiques, puisqu'elle n'emporte qu'une interdiction pour le représentant de l'État de déférer cette décision devant le tribunal administratif. Pour autant, elle n'est pas opposable aux tiers et n'emporte donc aucune garantie de l'État au profit de la collectivité. C'est la raison pour laquelle j'avais déposé un amendement visant à apporter aux collectivités une garantie de l'État

article 20. En matière d'urbanisme et d'autorisation d'occupation du sol, il est de jurisprudence constante que la responsabilité à rechercher est celle de la personne publique au nom de laquelle la décision fautive a été prise.

Un peu plus tard, la même commune demande une autre prise de position formelle aux services de la préfecture quant à l'opportunité de délivrer un permis de construire. Là encore, la préfecture, toujours la DDT, rend un avis formel positif sur la délivrance du permis, conforme au PLU élaboré et voté par la commune. Or ce permis, attaqué devant le tribunal administratif, est annulé. Le jugement est confirmé par la cour d'appel administrative, puis par le Conseil d'État. Des riverains sollicitent devant les juridictions civiles la démolition de la maison qui leur porte grief et obtiennent satisfaction. Le bénéficiaire du permis annulé et propriétaire de la maison démolie se retourne alors contre la commune qui lui a délivré le permis de construire après l'avis favorable donné par la préfecture. Il sollicite des dommages et intérêts dont le montant est égal à la valeur de la maison démolie.

François Bonhomme, sur l'article. Cet article vise à rendre opérationnelle une attente forte des élus locaux, et singulièrement des maires, celle d'un État qui accompagne les collectivités locales dans leurs tâches et dans l'exercice de leurs missions- missions- attente forte, très souvent annoncée, souvent avec ostentation, et pourtant très largement déçue. La création d'une procédure de rescrit, ou de demande de prise de position formelle, pour les collectivités locales, comme il en existe dans d'autres domaines, et ce pour des actes posant des questions de droit, me semble de nature à alléger, à fluidifier l'exercice des responsabilités et le travail quotidien des exécutifs locaux. Pour peu qu'un délai raisonnable soit retenu pour obtenir une réponse, cette procédure constituerait une amélioration significative pour le fonctionnement courant

Cela revient à donner une latitude nouvelle aux élus pour stabiliser et réduire certaines incertitudes et fragilités juridiques. J'ajoute que cela ouvre la voie à un renversement attendu en favorisant une logique de conseil plutôt qu'une situation de tutelle et de contrôle.

Leroy, vise à rendre obligatoire la prise de position formelle par le préfet en cas de saisine. Dans la mesure où la prise de position formelle exclut un déféré préfectoral, l'adoption conduirait à un report temporel de la charge de travail des services de l'État, puisque tous les actes des collectivités territoriales sont aujourd'hui transmis et analysés. S'il y a davantage de prises de position formelle, l'analyse des actes dans le cadre du contrôle de légalité sera allégée. Quel est l'avis de la commission

monsieur le ministre,

fallait peut-être transformer le corps préfectoral, et en particulier les services de contrôle de légalité, en conseil des collectivités, sans pour autant faire tomber le délai juridictionnel de deux mois ni le principe selon lequel le silence gardé

tenu de répondre dans un délai de deux mois. Si, à titre exceptionnel, il ne le fait pas, il en informe le maire en lui donnant les raisons de cette non-réponse.

Cet amendement s'inscrit dans le chapitre visant, selon l'expression du Gouvernement, à « fluidifier les relations entre l'État et les collectivités ». On l'a dit et répété, l'article 20 permet aux collectivités territoriales de saisir le représentant de l'État dans le département pour s'assurer de la légalité d'un projet d'acte soulevant un point de droit, sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le préfet en cas de circonstances nouvelles et sur les autres points de droit du même acte desquels il n'aurait pas été saisi. Cette saisine serait privée de tout effet par rapport aux situations particulières, complexes et irritantes actuelles, si la loi n'explicitait pas la source même de ces questions,

explicitement dans la loi l'état actuel de cette jurisprudence, afin que les préfets puissent disposer d'une source législative simple et claire, sans avoir à rechercher tous les éléments de jurisprudence ou de doctrine en la matière. Le dispositif proposé respecte scrupuleusement l'état du droit, tout en l'affirmant d'une façon non équivoque. Il lève ainsi les contradictions incessantes entre les angles d'interprétation des administrations centrales

les collectivités territoriales, en particulier les petites communes et leurs groupements, souvent isolés et sans service juridique, bénéficient du regard bienveillant de l'État dans les démarches et procédures qu'elles doivent accomplir. Dans l'hypothèse où une erreur de bonne foi pourrait être commise, dans le cadre strict prévu par le code des relations entre le public et l'administration, il pourrait être utile de faire bénéficier les élus du droit à l'erreur applicable à tous les administrés. La parole est à M.

la question du droit à l'erreur se pose aussi pour les collectivités locales, qui sont de plus en plus soumises à des risques d'erreur et, par là même, à des risques en termes de responsabilité,

L'Assemblée nationale ne l'avait pas maintenue, considérant que le projet de loi portait uniquement sur les entreprises et les particuliers, sans remettre en cause le bien-fondé d'un droit à l'erreur,

avait été institué en 2018 par la loi pour un État au service d'une société de confiance. En effet, la rédaction de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui évoque des « personnes », sans autre précision, ne paraît pas exclure les collectivités territoriales. Pour autant, nous ne

Cet amendement est issu d'un retour d'expérience personnel. La gestion de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen a montré les carences du système d'alerte et d'information aux populations,

derniers sont, au même titre que les préfets, chargés d'avertir et de protéger la population lorsqu'un risque imminent se présente. Afin de mettre en place dans les meilleures conditions et de façon efficace la palette d'outils mise à disposition par le SAIP, les maires doivent être tenus au courant en continu de l'évolution de la situation. Or, sur un certain nombre de points, l'autorité préfectorale exerce une compétence exclusive. Lors d'un événement grave, la population, le plus souvent, se tourne en premier lieu vers le maire. Il se peut alors que ce le maire. Il se peut alors que ce dernier se trouve injustement pris à partie pour sa mauvaise gestion des événements ou pour l'imprécision des réponses Cet amendement vise donc à ce que le préfet transmette sans délai les informations dont il dispose au maire, afin que celui-ci puisse exercer sans entrave les prérogatives qui sont les siennes dans le cadre du SAIP. Quel est l'avis de la commission ?

une parité entre les élus locaux, d'une part, et les représentants des différents organismes et de l'État, d'autre part. En effet, si les communes et les intercommunalités exercent la compétence en matière d'urbanisme, dans les faits, elles ont peu de poids dans les avis rendus par les CDPENAF. Créer une parité entre élus et organismes permettrait de combattre le sentiment d'impuissance des maires face à des décisions qui leur échappent, sans pour autant remettre en cause l'équilibre décisionnel des CDPENAF. Quel

que celle-ci nécessite une maîtrise des outils numériques, auxquels l'accès n'est pas égal à toutes et tous. Après l'intercommunalité à marche forcée, nous voilà confrontés à la dématérialisation à marche forcée. Si le Gouvernement souhaite aller dans cette voie, il faudrait permettre aux secrétaires de mairie, notamment, d'être formés à une telle évolution. Le développement de la dématérialisation des services publics,

comme l'a souligné le Défenseur des droits, Jacques Toubon, en estimant que la numérisation peut aussi créer une inégalité d'accès aux services publics. Il rappelle par exemple que 19 % des Français n'ont pas d'ordinateur à leur domicile, que 27 % d'entre eux n'ont pas de smartphone et que plus de 500 communes françaises sont dépourvues de toute connexion internet et mobile. La dématérialisation engagée aux motifs de développer le numérique et de faire des économies ne doit pas se faire sur le dos de l'accessibilité et de la qualité des services publics.

En l'état actuel du droit, ceux-ci sont élus parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des EPCI qu'ils représentent. Le caractère obligatoire de cette restriction légale à l'éligibilité ne nous semble pas justifié. Aussi est-il prévu d'ouvrir la faculté de se porter candidat à ces fonctions à d'autres acteurs : les conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux,

La loi du 17 mai 2011 et le décret du 27 février 2015 renvoient à un règlement départemental de défense extérieure des distances entre les points d'eau et les habitations. Or, d'un département à l'autre, ces distances sont très variables. Dans certains départements, les distances

Cet amendement vise à préciser que le représentant de l'État doit veiller à ce que les règles départementales relatives à la défense extérieure contre l'incendie ne conduisent pas à faire obstacle à un développement raisonnable et maîtrisé des communes. Le cas échéant, il s'efforce à ce que des mesures nécessaires pour remédier à cette situation

Lorsque ce quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance ou lorsqu'il cesse de l'être en cours de séance, le maire peut convoquer de nouveau le conseil municipal à trois jours francs au moins d'intervalle. À la suite de la deuxième convocation, la règle du quorum ne s'applique Or, surtout dans les petites communes, mais pas seulement, il est parfois compliqué d'obtenir ce quorum. Par ailleurs- nous l'avons tous constaté dans les assemblées que nous avons fréquentées -, il peut arriver que certains élus d'opposition fassent fassent usage de la règle du quorum pour nuire au bon fonctionnement de la municipalité. Je vous propose donc d'assouplir cette règle en ne la rendant obligatoire que pour les questions budgétaires. Le but est de simplifier le fonctionnement de nos assemblées, mais aussi et surtout de responsabiliser les élus, afin d'éviter certaines absences.

La séance est reprise.

confortée par la commission des lois qui va jusqu'à vouloir leur suppression ! Non ! Histoire de faire des économies, cet article balaye d'un même mouvement d'autres outils que sont les conseils pour les droits et devoirs des familles, les annexes de mairies et certains rapports. les conseils de développement sont obligatoires dans les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants et permettent d'approfondir la participation citoyenne. Pourtant, le Gouvernement souhaite les rendre facultatifs et restreindre leur pouvoir consultatif ! Pourtant, la majorité sénatoriale propose de les supprimer En octobre 2018, la ministre Jacqueline Gourault défendait la généralisation de ces instances, les préfets ayant même reçu une instruction sur ce sujet. Que s'est-il passé depuis ? Pourquoi proposer un tel recul au moment où les citoyens et les citoyennes sont de plus en plus demandeurs de démocratie participative, afin d'avoir une prise sur les décisions ? Envoyer de tels signaux négatifs ne pourra que conduire à freiner l'essor des conseils de développement, qui permettent pourtant d'intégrer des personnes bénévoles à la vie locale. Ces femmes et ces hommes ne demandent qu'à donner de leur temps pour partager leurs compétences personnelles au profit de la communauté. Pourquoi ne pas encourager un tel engouement pour la, la chose publique, dont le fonctionnement s'enrichit de la diversité des débats ? Quel est

adaptée à leur territoire. Nous avons réintroduit, dans le pacte de gouvernance, un certain nombre d'éléments. En raison de l'objet même du texte que nous discutons,

Rendre facultatifs ces conseils dès maintenant briserait l'élan et constituerait un retour en arrière en matière de mobilisation citoyenne, en fragilisant les plus récents d'entre eux, dans un contexte de renouvellement des mandats. Il apparaît donc que le projet de loi ne prend pas en compte les apports des conseils de développement. Outre leur contribution à l'enrichissement des politiques publiques, ils constituent, à l'échelle intercommunale, l'un des seuls lieux organisés dans lesquels les désaccords peuvent s'exprimer de manière argumentée et se résorber de façon apaisée. Dans un contexte marqué par la défiance et l'urgence écologique, ils font vivre et contribuent à diffuser les valeurs d'écoute et de respect de l'autre, d'attention à l'intérêt général et d'une citoyenneté active et responsable. Il est donc nécessaire de conserver l'article L. 5211-10-1 dans sa rédaction actuelle et de réaliser une évaluation permettant de définir, en connaissance de cause, les évolutions à apporter aux conseils de développement.

crise démocratique et de confiance entre les citoyens et les élus, monsieur le ministre, vous envisagez de rendre facultatif le seul dispositif participatif qui rapproche les élus intercommunaux, naturellement éloignés de nos concitoyens,

des gens qui n'ont pas d'autre latitude pour s'exprimer que celle-ci. Il existe de nombreuses expériences réussies de conseils de développement. Je pense, par exemple, à celui de Nantes. Il est vrai, d'autres conseils de développement

C'est l'histoire récente de notre vie politique : le débat démocratique, notamment au moment du grand débat, a été très nourri sur cette demande de proximité et d'échanges avec

d'autant que celui de Bordeaux fonctionne très bien. Monsieur le ministre, c'est le conseil de développement qui a mené de façon très efficace le grand débat

par la loi NOTRe en 2015, les conseils de développement sont des outils de démocratie participative, de dialogue et de consultation. Chaque conseil de développement est libre de s'organiser comme il le souhaite. Cette souplesse permet une application adaptée aux particularités territoriales de chaque EPCI.

métropoles ou des communautés urbaines où le besoin de démocratie participative est souvent le plus prégnant. L'amendement

sur la transparence des mutualisations en cours. En supprimant les schémas, nous supprimons également l'obligation de faire un point d'étape annuel. La Henri Cabanel, pour présenter l'amendement n° 214 rectifié. Cet amendement vise à maintenir l'article L. 5211-39-1 du code général des collectivités locales, qui prévoit que le président de l'EPCI à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'EPCI et ceux des communes membres. Ce rapport comporte notamment un projet de schéma

participative n'est ni détruite ni niée par le travail de la commission des lois. Soyons précis et factuels : nous n'interdisons pas et nous ne supprimons pas

de la Coordination nationale des conseils de développement. Je lui ai indiqué que nous reconnaissions la valeur de toutes les instances de démocratie participative. Quoi qu'il en soit, nous ne tenons pas notre légitimité de droit divin ou de droit républicain

dans le pacte de gouvernance, la possibilité pour les intercommunalités de définir comme elles le souhaitent leur mode d'association et de consultation des acteurs de la société civile. Il me semble que nous avons donc

l'aventure. Rares sont les communes de taille significative aujourd'hui qui contourneraient le principe même d'un conseil de quartier. Tout simplement parce que nous sommes des élus

pouvoir d'autosaisine. Bref, non seulement vous les rendez facultatives, mais vous les ravalez au rang de simples comités consultatifs. Monsieur le ministre, vous nous dites qu'en

Dans les communes ou EPCI de plus de 100 000 habitants, dans les départements et les régions, ces frais peuvent atteindre des montants importants, difficilement contrôlables. Pour plus de transparence,

Dans ce cadre, il est notamment prévu que le médiateur territorial transmette chaque année un rapport d'activité pouvant contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou du groupement considéré. Au-delà, je propose que ce rapport fasse l'objet d'un débat au sein de l'organe délibérant.

qui constituent un patrimoine non protégé, mais qui doit absolument être sauvegardé, ce que ne peuvent pas toujours se permettre les plus petites communes. C'est pourquoi le groupe du RDSE est très favorable à cet article 24, lequel étend à toutes les opérations d'investissement du bloc communal la faculté pour le préfet d'accorder une dérogation

Concernant les projets d'investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, cette participation minimale du maître d'ouvrage peut déjà faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de l'État dans le département. Cet amendement a uniquement pour objet de fluidifier la procédure d'autorisation de cette dérogation en cas de catastrophe naturelle, en tendant à considérer que l'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle dans le département où se situe le projet d'investissement fait office d'autorisation préfectorale.

Peut-être faut-il donc réfléchir à étendre cette dérogation, dans des périmètres très précis, au-delà des petites communes, car le patrimoine ne connaît pas de limites de population.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

était circonscrite au patrimoine non protégé en péril, mais, compte tenu des problèmes de financement rencontrés par les collectivités et les maîtres d'ouvrage, y compris

par nombre de mes collègues. La loi prévoit une obligation, pour les propriétaires, d'entretien de la façade des immeubles à Paris et dans un certain nombre de villes françaises : dans ces communes, « les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.

Cette mesure permettrait de soutenir les efforts de revitalisation des centres-bourgs effectués par les communes et d'éviter, par exemple, qu'un bâtiment délabré ne nuise à l'attractivité d'une commune et à son cadre de vie. Les règles en matière d'entretien des immeubles sont aujourd'hui insatisfaisantes ; le pouvoir des communes relève davantage des normes d'urbanisme, dont le respect est notamment

le propriétaire à réaliser les travaux d'entretien ; en cas de non-réalisation dans les six mois, il peut prendre un arrêté en vue de les prescrire ; si les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti, il peut peut les faire exécuter d'office, à la charge du propriétaire, avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance, ce qui garantit le respect du droit de propriété, si important dans notre pays.

délier les services de l'État, sans motif d'intérêt général suffisant, de secrets protégés par la loi, comme le secret fiscal, mais aussi des obligations imposées aux responsables du traitement des données personnelles par le droit européen, à travers le règlement général

sont contraires au premier alinéa de l'article 38 de la Constitution. En conséquence, la présente motion tend à proposer au Sénat de déclarer ces amendements irrecevables en application de l'article 44 ,

du maire, c'est-à-dire autre chose que la simple amélioration des conditions d'exercice du mandat, aussi importante soit-elle, la mort tragique du maire de Signes, dans le Var, en tentant de faire appliquer la loi municipale, m'en aurait définitivement convaincu. Pas de sécurité des élus chargés de faire respecter la règle commune sans reconnaissance publique de la dignité d'une fonction exercée au nom de la collectivité, souvent même au nom de l'État une fonction qui n'est pas un passe-temps honorifique pour désoeuvrés fortunés, qui pourraient donc se passer d'indemnités, mais la condition de possibilité de la République territoriale. L'institution d'un statut de l'élu communal serait le signe de cette reconnaissance et chacun sait dans cet hémicycle qu'en la matière les symboles comptent.

prévu, se sont aperçus que le maigre pécule avec lequel ils avaient quitté leur département était épuisé. Afin de permettre à la démocratie de fonctionner, on a ainsi inventé l'indemnité pour compenser un manque à gagner. La

de la monarchie de Juillet auraient pu siéger au Parlement. Tous ceux qui sont profondément attachés à cette épopée républicaine, qui a vu des citoyens français abandonner leur métier pour devenir des représentants de la Nation ou, plus tard, des maires, des conseillers généraux, puis départementaux, sont sensibles à cette idée : il faut maintenir ce principe, tout en veillant à ce qu'une juste indemnité permette- de manière forfaitaire, hélas ! -de compenser les pertes

avec ces amendements, il faut continuer à y répondre en marquant notre attachement à la notion de gratuité, corollaire du service qui est rendu par l'élu à ses concitoyens. C'est la raison pour laquelle, après en avoir délibéré plusieurs fois, parce qu'il s'agit d'une position constante de la commission, nous avons souhaité maintenir ces principes, tout en étant attentifs à améliorer la situation matérielle des

C'est une richesse pour la collectivité territoriale qui en bénéficie. Une politique active de valorisation de ces talents à l'issue du mandat électif serait de nature à rajeunir les conseils des collectivités territoriales. Il s'agit non seulement d'inciter de jeunes actifs à détenir un mandat, mais aussi à s'investir pleinement dans la vie publique. Si les collectivités bénéficient grandement de l'expérience de la vie en société et du monde du travail tout aussi souhaitable que la société et le monde du travail bénéficient du sens de l'intérêt général et de la citoyenneté acquis à l'occasion de l'exercice de mandats électifs publics.

Il est proposé de relever le plafond indemnitaire que le conseil municipal peut décider d'allouer au maire ou aux adjoints des communes de moins de 3 500 habitants en créant une strate indemnitaire unique,

pour permettre de relever ce plafond et se rémunérer à la hauteur de leur engagement. Aussi, afin que cette mesure puisse véritablement être mise en oeuvre et ne reste pas un voeu pieux

Plus les EPCI sont grands, plus les collectivités sont grandes, plus ce temps de travail s'accroît. Un maire sur deux et un adjoint sur trois consacrent plus de 35 heures par semaine à leur mandat. Si les retraités sont 62 % à faire plus de 25 heures, seulement un tiers des actifs

comme le préconisait déjà le rapport Mauroy de 2000, un statut d'agent civique territorial qui correspondrait mieux à la réalité et permettrait, en outre, d'accroître la démocratisation

Qui croyons-nous berner en refusant inlassablement cette obligation que les citoyens réclament, certains étant d'ailleurs persuadés qu'elle existe déjà ? Quand arrêterons-nous d'être décalés à ce point de la réalité ? De quoi avons-nous peur ?

Faire reconnaître le droit des élus pour développer l'engagement est une nécessité dans le contexte politique de défiance actuelle. Un État démocrate a pour souverain le peuple, comme le dispose l'article 3 de la Constitution. Ce peuple souverain s'éloigne des urnes, renie les partis traditionnels et réclame des mesures qui dérangent et déstabilisent notre petit monde : reconnaissance du vote blanc, obligation du casier vierge. Au mieux pudiquement, au pire agressivement, les élus nationaux parlent de démagogie et actent comme seul blanc-seing les scrutins. Mais quel pourcentage d'abstention ou de votes extrêmes provoquera un électrochoc de raison ? Mon amendement visait simplement à rétablir une équité. Je rappelle inlassablement dans cet hémicycle que près de 400 professions exigent de leurs candidats qu'ils aient des casiers vierges.

l'esprit reste le même, à savoir la recherche de l'exemplarité de l'élu dès sa candidature.

l'extension du bénéfice du congé pour la campagne électorale, tel que le prévoit le code du travail, aux salariés qui seraient candidats dans les communes de moins de 1 000 habitants. C'est une bonne chose. Il est cependant muet sur la situation qui prévaudra

Pour respecter le travail de la Haute Assemblée, encore faudrait-il daigner lui répondre quand, courrier après courrier, nous sollicitons, non pas des réponses fermes, mais simplement des avis.

aux adjoints et conseillers exerçant la fonction de président ou de vice-président des syndicats de communes. Alors même que leurs fonctions nécessitent un engagement supplémentaire, certains de ces adjoints et conseillers ne bénéficient guère de cette majoration pourtant nécessaire pour assurer l'administration de la commune. Un article du code général des

des raisons diverses et variées, à commencer par l'élargissement des périmètres intercommunaux. Toutefois, des dispositifs existent déjà : les membres des exécutifs locaux peuvent demander à suspendre leur contrat de travail,

que les élus puissent exercer leur mandat sans que cela leur coûte personnellement et professionnellement. Dans cette perspective, le présent amendement tend à ce que le temps du mandat, en cas de suspension du temps de travail, soit pris en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.

Cet amendement nous semble très important, car il a pour objet de faire bénéficier les maires et leurs adjoints du statut de salarié protégé. Le dernier alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà que ces élus « sont sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. » Cependant, ce renvoi global à cette division du code du travail rend cette protection inopérante, le livre IV compte une multitude de cas et de procédures, sans que l'on sache exactement laquelle ou lesquelles s'appliquent effectivement aux salariés titulaires d'un mandat électif. Il est donc indispensable d'intégrer au sein du code du travail des divisions spécifiques concernant le cas des salariés titulaires d'un mandat électif et d'y préciser les procédures qui leur sont applicables. En l'espèce, l'amendement tend à ce que le licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat électif ne puisse intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et à ce que cette autorisation soit également requise durant les douze mois suivant l'expiration du mandat du salarié. Lorsque le ministre compétent annule, exerçant ainsi son recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement, ou lorsque le juge administratif annule la décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié a le droit d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

électif pour garantir leur statut de salarié protégé, le présent amendement tend à préciser les règles qui leur sont applicables. Le renvoi global au livre IV de la deuxième partie du code du travail étant insatisfaisant, il faudrait préciser que ce sont les règles relatives aux délégués syndicaux et anciens délégués syndicaux qui leur sont applicables. Ainsi, l'article 26 serait satisfait,

entre, d'un côté, la protection garantie par le droit du travail dans l'entreprise et, de l'autre, une fonction élective issue du suffrage. Je n'ouvrirai pas un débat que je ne saurais pas refermer, mais la question pourrait aussi se poser pour les élus consulaires, comme les

que nous sommes en train de soulever des questions juridiques et des questions de principe dont nous devons bien mesurer la portée. D'abord, il est vrai que les principes fondamentaux du code du travail impliquent la protection d'un

protéger, puisqu'elle l'est aussi afin de favoriser le dialogue social dans l'entreprise et de faire en sorte que ce dialogue social s'accomplisse de bonne foi. C'est pour cette raison d'ailleurs que la charge

Mais à partir du moment où l'on applique les mêmes protections à des salariés qui exercent des activités qui ne sont pas au service de l'entreprise, se pose vraiment une question de principe. Je ne veux pas y répondre définitivement maintenant, car je crois que le débat mérite d'avoir lieu, mais ce que je relève après avoir écouté le ministre, c'est que ce débat n'est pas simple à trancher. Il ne peut pas l'être dans la précipitation. Par ailleurs, je ne me sens pas totalement légitime, en tant que président de la commission des lois, d'empiéter ainsi sur les attributions de la commission des affaires sociales, qui est la gardienne des principes fondamentaux du code du travail.

Je voterai contre ces amendements, et je souhaite que la navette nous permette de trouver une solution qui ne soulèvera pas les objections que je redoute, parmi lesquelles celle qu'a exposée le ministre à l'instant sur le fait que, à force de vouloir protéger les élus vis-à-vis de leur employeur, on risque tout simplement d'atteindre le résultat exactement inverse

même mieux que moi, les employeurs ne sont pas forcément des multinationales : c'est l'entreprise du bâtiment, la petite entreprise de travaux publics, quand ce n'est pas le charcutier traiteur.

dans l'hémicycle est de nature à nous éclairer davantage que les débats très rapides que nous avons pu mener sur le sujet en commission.

La parole est à M. Loïc Hervé, pour explication de vote.